Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quel contexte abordons nous ce débat proposé par notre groupe ? un Français sur cinq est touché par des problèmes de santé mentale, soit près de 13 millions de personnes, et 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Les Français sont ceux qui consomment le plus d’anxiolytiques au monde. À l’occasion du Congrès français de psychiatrie et psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent en 2023, les professionnels ont constaté que

un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge indique que la consommation de médicaments visant à soigner la santé mentale a doublé chez les 6 17 ans. Faute de prise en charge adaptée, les prescriptions de médicaments psychotropes ont explosé et 5 % de la population pédiatrique, c’est à dire des bébés et des tout petits, se voient même prescrire des psychotropes.

Le coût économique et humain direct et indirect des problèmes de santé mentale est évalué à 110 milliards d’euros. C’est fort de ces constats et de ces chiffres, qui ont de quoi donner le vertige, que, le 10 octobre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le Premier ministre Michel Barnier érigeait la santé mentale grande cause nationale

le nombre de passages aux urgences pour geste suicidaire chez les enfants de 11 à 17 ans, qui avait augmenté de 70 % au milieu des années 2020, a fortement baissé. Les tensions aux urgences étant moindres, ce service public de première ligne a repris force et vigueur et n’est plus contraint de réguler ses accès.

bénéficiaient d’une prise en charge spécialisée, en 2040, toute une génération obtient une réponse acceptable, dans des délais suffisamment courts pour que les soins soient pertinents et les effets tangibles. Et les jeunes parents,

en ouvrant 15 000 postes de psychologue dans l’éducation nationale ; en déployant un programme massif, et surtout continu, de formation de la communauté éducative ; en développant les bureaux d’aide psychologique universitaire.

les territoires ? En consolidant et en finançant suffisamment les CLSM et les projets territoriaux de santé mentale, et en mettant au cœur de l’offre de soins les droits des usagers et des aidants.

d’où que l’on vienne, qui que l’on soit. Je veux croire que, ici, nous pouvons prendre ensemble des décisions de long terme qui changeront radicalement la situation de la santé mentale et donc la vie des Français. Cette ambition, je sais que nous la partageons tous ici. Jaurès, « le courage, […] c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ». Je ne méconnais pas la réalité budgétaire qui est la nôtre, en 2025, mais je sais que nous devons voir loin pour les politiques de prévention, notamment en santé mentale ; nous devons prévenir pour arrêter de mal guérir. Pour arriver à cet idéal, pour relever ce défi, il nous faut de la constance et du sérieux. Or, de la constance, nous n’en manquons pas au Sénat, et du sérieux non plus. Combien de rapports – j’attends avec impatience celui de mes collègues de la commission des affaires sociales – ont déjà tracé les contours de ce que nous devons faire,

ans à la santé mentale doit être actée et appliquée avec rigueur. Sur le modèle de la loi de programmation militaire, qui a pour vocation de faire de la France une puissance d’équilibre et de garantir les moyens alloués à notre sécurité, une telle loi permettrait de faire de la France un pays où nos concitoyens retrouvent l’équilibre et la sécurité structurelle Je sais que cette ambition pragmatique dépasse largement les clivages politiques. La santé mentale des Français serait gagnante, les finances publiques le seraient aussi. Faisons le pari ensemble de l’optimisme pour parvenir à la France de 2040 que je vous ai décrite

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, la santé mentale est l’un des grands défis de notre

publiquement. En effet, je partage tout à fait l’ambition autour de laquelle nous nous réunissons ce soir : celle de nous donner les moyens de faire de cette grande cause qu’est la santé mentale une priorité. se demander comment nous donner les moyens d’en faire une cause durable, car l’état inquiétant de la santé mentale de nos concitoyens, notamment d’une partie de notre jeunesse, nous oblige

Les besoins de soins ne cessent d’augmenter, révélant à la fois une meilleure acceptation des troubles psychiques et la nécessité d’adapter notre système de santé. En parallèle, les professionnels font face à des tensions croissantes : attractivité en berne, surcharge de travail ou encore manque de ressource médicale. Nous sommes tous concernés par ce qui représente un enjeu prioritaire de santé, indissociable de la santé globale, mais qui est aussi, plus largement, une véritable question de société. Dans ce contexte, nous devons avoir un cap commun : faire en sorte que cette grande cause soit non pas un slogan ou un phénomène éphémère, mais un mouvement de fond.

qui fait directement écho à notre débat de ce soir. C’est d’ailleurs votre assemblée qui, la première, avait érigée la santé mentale, et spécifiquement celle des jeunes, en grande cause de dimension nationale, en janvier 2024, avec une résolution votée sur l’initiative de la sénatrice Nathalie Delattre. Cet engagement parlementaire fait écho à des mentalités qui évoluent. On parle de plus en plus, et de plus en plus librement, de santé mentale dans les écoles,

Dans cette perspective et en lien avec le Parlement, la responsabilité du Gouvernement, et du ministre de la santé en particulier, est d’ancrer notre politique en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie dans une ambition de long terme, clairement affirmée et transversale.

interministériel. J’ai pu, à cette occasion, insister sur mes priorités d’action, que je vais décliner devant vous. La première priorité est le développement de l’accès aux soins et le renforcement de la prévention.

autant de dispositifs qui prennent de l’ampleur et que je veux renforcer pour garantir un accès rapide aux soins psychologiques et psychiatriques. J’entends aussi poursuivre et amplifier la montée en charge de Mon soutien psy, qui, je le rappelle, est accessible et remboursé dès l’âge de 3 ans.

Je vous réaffirme par ailleurs mon souhait d’engager une réforme des urgences psychiatriques, afin de garantir une prise en charge adaptée dans chaque territoire et de désengorger les services hospitaliers, à la suite du rapport parlementaire qui m’a été récemment remis par les députées Sandrine Rousseau et Nicole Dubré Chirat. Vous le voyez, je compte bien m’appuyer sur les nombreux travaux parlementaires. Toujours dans cette logique de mobilisation collective et transversale, j’ai demandé hier à la Commission nationale de la psychiatrie d’élaborer des propositions d’évolution de la psychiatrie de de secteur pour qu’elle puisse, d’une part, mieux se coordonner avec les autres dispositifs du paysage psychiatrique comme les centres experts et, d’autre part, réduire les délais de prise en charge en centre médico psychologique, qui sont souvent encore trop longs.

nous allons renforcer les maisons des adolescents et les CMP infanto juvéniles afin de répondre à la détresse psychologique croissante des enfants et des adolescents, tout en permettant une meilleure orientation dans l’offre de soins existante. Nous allons aussi porter une attention spécifique aux plus vulnérables, notamment aux enfants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et aux familles les plus précaires. Je veux également insister sur l’importance que j’accorde à la lutte contre toutes les formes d’addiction, une source importante de souffrance psychique, qu’elles qu’en soient les causes et les conséquences aggravantes.

en particulier permettre à plus d’étudiants en santé d’effectuer un stage en psychiatrie pendant leur cursus. Il en ira de même pour le cursus paramédical des infirmiers. Cela leur permettra de découvrir très concrètement cet univers plus tôt dans leurs études, alors que 37 % des futurs médecins avouent encore que la psychiatrie continue de leur « faire peur ». Je sais que cette appréhension vis à vis de la psychiatrie s’explique en partie par plusieurs drames, y compris très récents, liés à des actes de violence commis par des patients relevant de la psychiatrie.

en matière de sécurité dans les établissements psychiatriques. Ce rapport évoquait le nombre de 10 000 fugues par an chez les patients hospitalisés sans consentement, ainsi qu’une vingtaine d’homicides sur cinq ans. Il dénonçait une sous estimation des agressions, notamment sexuelles, et une organisation sectorielle peu adaptée à la diversité des pathologies. Or des drames récents prouvent que des failles demeurent. Il y a quinze jours, à Massy, dans l’Essonne, département dont je suis élue, une femme a perdu la vie, poussée sur les rails du RER B par un homme souffrant de troubles psychiatriques et ayant fugué d’un établissement spécialisé. Je veux le dire avec force : il ne s’agit pas de stigmatiser les personnes malades, elles mêmes victimes de leurs propres troubles, ni de mettre en cause les soignants, qui ne sont ni gardiens de prison ni agents de sécurité. Toutefois, il nous incombe de viser ensemble deux objectifs fondamentaux garantir les droits et la dignité des personnes hospitalisées sans leur consentement, tout en ne renonçant pas à la sécurité de tous. Cet homicide, comme d’autres, nous impose une feuille de route claire pour sécuriser les établissements, prévenir les fugues et protéger patients, personnel, familles et citoyens. C’était en partie l’enjeu du plan pour la sécurité des professionnels de santé publié en septembre 2023 qui, parmi quarante deux mesures, prévoyait notamment d’améliorer la formation,

d’un grand pas en avant pour nos concitoyens, qui nous amène à nous poser la question de l’effectivité de la prise en charge des patients en France et de l’adaptation de notre système de santé à la prise en compte d’un phénomène qui est de moins en moins ignoré.

les services ne peuvent plus fonctionner pour aider nos plus jeunes. Ce sont ainsi 2 500 enfants et jeunes qui se retrouvent sans solution, sur un bassin de vie de 240 000 habitants. Or, si les troubles ne sont pas traités au plus tôt, les pathologies psychiatriques vont se cristalliser et être encore plus difficiles à traiter. Nous considérons que le système de santé et de protection sociale doit s’appuyer sur le triptyque accompagnement traitement soins adaptés pour chaque patient.

dans plusieurs champs, notamment les dépressions résistantes, les troubles bipolaires, la schizophrénie et l’autisme de haut niveau, avec des pratiques harmonisées et un référencement

80 % de ces médicaments sont prescrits par des médecins généralistes, parfois sans suivi psychologique et médical adapté, malgré les graves risques de dépendance et d’effets secondaires. On estime que 20 % seulement des patients suivent une psychothérapie parallèlement

À quand une orientation systématique des patients sous psychotropes vers un professionnel de santé mentale et une psychothérapie ? À quand une généralisation sans discrimination du remboursement des séances de psychothérapie pour l’ensemble de la population, y compris en cas de troubles sévères, de risques suicidaires, de

Elles sont souvent marginalisées et vivent dans une grande précarité dans nos communes. À ce jour, 75 % des personnes sans abri présentent des troubles psychiatriques en raison de parcours complexes, de problèmes de santé mentale non détectés et non suivis. Leur accès aux soins est problématique : le manque d’accessibilité tant géographique que financière les éloigne d’une offre de soins adaptée. Les services de psychiatrie sont saturés et peinent à recruter. Les professionnels spécialisés manquent cruellement et les soignants généralistes ne sont pas formés, des troubles de la santé mentale. Ces difficultés de prise en charge se répercutent sur le quotidien des maires, démunis face aux troubles à l’ordre public provoqués par des personnes laissées sans solution. Je pense par exemple au maire de Saint Brieuc, agressé physiquement par un homme laissé sans suivi après des prises en charge ponctuelles, et connu des services médicaux, sociaux et de sécurité de la ville.

que comptez vous faire pour que ceux qui sont déjà éprouvés dans leur quotidien par des accidents de la vie soient mieux accompagnés face à leurs problèmes de santé mentale ? Quels investissements envisagez vous pour développer l’« aller vers » et soutenir les maires démunis ? Comment rendre les métiers de la santé mentale attractifs pour les psychiatres,

Je pense notamment aux médecins et aux infirmières scolaires. Sur 1 800 postes budgétés en médecine scolaire, seuls 650 sont effectivement pourvus. Et 200 d’entre eux le sont par des contractuels. C’est bien trop peu pour être efficace

sur l’état des lieux de la santé mentale depuis la fin de la crise sanitaire. Nos travaux ont confirmé ce que chacun de nous observe dans son département : les centres médico psychologiques sont à bout de souffle. Alors qu’ils sont conçus comme le pivot de la prise en charge des troubles psychiques, le délai d’attente moyen pour une première consultation

nous ont fait part de leurs difficultés à obtenir des moyens pour leur CMP. Les agences régionales de santé (ARS) accordent en priorité des financements aux organisations particulièrement innovantes. Ces centres ne sont pas toujours innovants,

au moins accorder des crédits à des postes d’infirmiers en psychiatrie et d’infirmiers en pratique avancée

En témoignent les résultats de l’enquête nationale en collège et en lycée menée par l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec le ministère

présentent un risque important de dépression ; 24 % des lycéens déclarent qu’ils ont eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois ; 13 % d’entre eux indiquent avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie, sachant que 3 % de ces tentatives ont entraîné une hospitalisation. La pandémie de la covid 19 et les confinements successifs ont sans doute aggravé la santé mentale de nos jeunes. Le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, Frank Bellivier, soulignait le 26 mars dernier devant la commission des affaires sociales du Sénat que, depuis la crise sanitaire, il ne constatait « pas de dégradation, [que] la situation ne s’amélior[ait] pas non plus : les indicateurs d’anxiété, de dépression, de troubles du sommeil et d’addiction restent relativement élevés, en particulier chez les jeunes ». Face à une jeunesse en perte de repères et inquiète pour son avenir, je m’interroge sur le rôle et les moyens de l’école, un lieu de passage obligé, qui peut être celui de l’épanouissement comme celui du harcèlement. Et même si l’école ne peut pas tout, elle pèse pour beaucoup dans la construction de la personnalité d’un élève. Alors, monsieur le ministre, comment l’école pourrait elle devenir davantage un lieu de prévention et de sensibilisation aux enjeux liés à la santé mentale ? Au delà des numéros d’urgence, du protocole de santé mentale dans chaque établissement et de la démarche École promotrice de santé, qui peuvent être des outils efficaces,

Troubles du sommeil, anxiété, isolement, décrochage, les difficultés sont nombreuses et s’accentuent face à la pression académique et aux incertitudes liées à l’avenir.

Des dispositifs existent, mais ils doivent être renforcés et mieux intégrés aux parcours des jeunes. Certes, la reconnaissance de la santé mentale comme grande cause nationale pour 2025 est une avancée importante, que je salue. Je souhaite à ce titre rappeler l’engagement de notre ancienne collègue Nathalie Delattre, notamment au travers de sa proposition de résolution visant à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale, adoptée ici même à l’unanimité. Mais il faut aller plus loin en augmentant le nombre de psychologues dans les universités, en sensibilisant étudiants et enseignants à la santé mentale, et en garantissant un accès rapide à des soins adaptés. Ma question est simple, monsieur le ministre : quelles mesures envisagez vous de prendre pour faciliter l’accès des étudiants à un accompagnement psychologique au sein même de leur établissement ?

L’éloignement géographique allonge en effet les temps de déplacement et freine l’accès à des droits fondamentaux tels que la santé ou l’emploi. L’isolement pèse aussi sur la santé mentale des jeunes ruraux. L’Igas note que les politiques en faveur de la jeunesse ont « élargi leur champ d’attention aux transitions de la jeunesse et aux inégalités », mais observe également que « les dispositifs plus spécialisés de formation, d’accompagnement vers l’emploi ou de santé […] se concentrent quant à eux dans des agglomérations plus importantes

garde toute sa vie un fonctionnement différent, avec une façon particulière d’agir, de penser ou d’entrer en relation avec les autres. Cela représente autant de défis à relever pour préserver sa santé mentale.

de la mission d’information sur les troubles du neurodéveloppement, qui nous a conduits à souligner le retard pris par la France en matière de diagnostic, mais aussi de prise en charge des TND. Ce retard est dû à un manque criant de psychiatres, de psychomotriciens, d’ergothérapeutes ou encore d’orthophonistes. d’information ont été reprises dans la proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants.

la décision si salutaire de Michel Barnier de faire de la santé mentale la grande cause nationale de 2025. La santé mentale des jeunes est préoccupante, tout comme le silence assourdissant qui règne tant dans le débat public que dans les politiques de santé publique sur l’un des leviers les plus insidieux de cette dégradation : la consommation de cannabis. Les Les autorités sanitaires doivent briser le tabou et montrer que le cannabis altère profondément les fonctions cérébrales en formation. Il ralentit la maturation du cerveau, dégrade la mémoire de travail et entrave les capacités d’apprentissage. Chaque jeune qui aspire à être libre – ce qui est heureux – devrait savoir que le cannabis affecte la manière même dont l’information est traitée. Le cerveau devient moins apte à trier, à hiérarchiser, à prendre du recul. Dans un monde saturé de contenus numériques, avec leur lot de fausses informations et autres manipulations destinées à propager des thèses très dangereuses, cette fragilité cognitive rend le jeune cerveau plus vulnérable aux influences les plus nocives. Le cannabis que l’on consomme pour être moins stressé empêche de gérer le stress, affaiblit la résilience face à l’effort, provoque une anxiété diffuse et mine la motivation.

Derrière chaque statistique, il y a une vie brisée par une substance que certains continuent de présenter comme inoffensive. Monsieur le ministre, que comptez vous faire, dans le cadre des campagnes de communication de la grande cause nationale, pour mettre un terme à cette illusion dangereuse d’un cannabis sans conséquence aucune pour la santé mentale ? Bravo ! La parole

Nous le voyons bien au travers des diverses interventions, la question de la santé mentale n’est plus une bombe à retardement ; elle est désormais une bombe à fragmentation, dont les dépressurisations psychologiques se sont multipliées à la faveur de la crise sanitaire, qui a agi comme un accélérateur ou un amplificateur.

de psychiatre à l’hôpital public sont vacants. Si les causes sont diverses, les professionnels évoquent avec insistance la question de la responsabilité juridique. Quelle réponse pouvez vous leur apporter ?

En effet, un Français sur quatre sera concerné par un trouble mental au cours de sa vie. Cette grande cause nationale s’articule autour de quatre objectifs prioritaires : la déstigmatisation le développement de la prévention et du repérage précoce ; l’amélioration de l’accès aux soins partout sur le territoire français ; et l’accompagnement des personnes concernées. Ces objectifs sont non seulement louables, mais indispensables. Il convient néanmoins de ne pas rester dans l’affichage et de les traduire par des actions concrètes.

pour repérer les troubles, pour financer des postes, notamment d’IPA, d’assistants médicaux ou de coordonnateurs au sein des établissements, mais également pour sensibiliser les équipes de professionnels accueillant du public. La création de maisons des enfants,

Dire que le sujet est d’importance est un euphémisme : plus de 12 millions de Français souffrent de troubles psychiques et une tentative de suicide a lieu toutes les trois minutes… Si la santé mentale a été désignée grande cause nationale, ce n’est malheureusement pas sans raison.

Avec plus de 23 milliards d’euros annuels, les dépenses remboursées au titre de la souffrance psychique et des maladies psychiatriques représentent le premier poste budgétaire de l’assurance maladie. En 2021, les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont souligné la nécessité d’une approche holistique, articulée aux besoins des territoires. Les structures locales – centres médico psychologiques, hôpitaux de proximité ou encore associations de santé mentale – jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des patients, au plus près des réalités du terrain. Leurs équipes connaissent mieux que quiconque les besoins spécifiques des communautés les élus locaux ont une responsabilité particulière. Ils sont les garants de la cohésion, du lien social et de la qualité de vie dans leur territoire. Ils ont le pouvoir d’impulser des dynamiques locales de mobiliser les acteurs de santé. Ils peuvent plaider pour des moyens supplémentaires auprès des instances nationales, ce que nous faisons à notre tour ce soir. Ce constat sanitaire appelle une meilleure articulation entre politique globale et déclinaisons territoriales. Ne serait il donc pas envisageable

dispose des moyens nécessaires pour répondre aux défis de la santé mentale.

santé, 13 millions de Français présentent un trouble psychique. Plus d’un quart de la population française consomme aujourd’hui des anxiolytiques, antidépresseurs et autres médicaments psychotropes. Les troubles psychiques sont ainsi la première cause d’invalidité, la deuxième cause d’arrêt de maladie et, avec 23 milliards d’euros en 2023, le premier poste de dépenses du régime général de l’assurance maladie. Ces chiffres doivent nous alerter, d’autant plus que la forte dégradation de la santé mentale depuis le covid 19 et les confinements successifs frappe sans distinction de milieu social ou d’âge. Il est urgent de repenser notre approche de la santé mentale : cette dernière est aussi importante que la santé physique. Je me réjouis donc que, dès octobre dernier, le Gouvernement ait fait d’elle la grande cause nationale de 2025. Véritable enjeu de santé publique, la santé mentale est l’affaire de tous.

Le manque de ressources adaptées pour les enfants présentant des besoins spécifiques, les délais d’attente dans les centres médico psychologiques ou encore les limites du dispositif Mon soutien psy l’illustrent : l’accès aux soins en santé mentale reste très dégradé.

la souffrance psychosociale ordinaire jusqu’aux maladies psychiques avérées, parmi lesquelles la dépression, les psychoses, les troubles liés à l’anxiété, les addictions, les tendances suicidaires, les psychotraumatismes et les troubles autistiques.

sont pris en charge par les services psychiatriques. Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 25 % des causes d’invalidité en France.

Ce dispositif, tourné vers le secteur libéral, ne saurait compenser les défaillances observées dans le secteur public. La fragilisation de la santé mentale touche davantage les femmes. Selon une étude de l’OMS,

l’administration publique, la filière de l’hébergement et de la restauration, l’hébergement médico social et l’action sociale. La santé mentale est le parent pauvre de notre système de santé. Depuis des décennies,

insuffisance de l’offre de formation et vieillissement des professionnels en activité. Or, depuis 2017, ni le Président de la République ni ses gouvernements successifs n’ont mesuré l’urgence d’agir pour reconstruire notre système de santé mentale ; deux feuilles de route ont certes été publiées,

est un facteur aggravant de la souffrance. Il est primordial de mener une réflexion globale et de travailler à une approche pluriannuelle de la santé mentale, un projet de loi de programmation prix réfléchir à un autre accompagnement de la souffrance mentale, par des institutions parfaitement adaptées à l’accueil des malades. Nous en